en précisant que ces dispositions portent également sur les différents organismes inter-établissements du réseau des chambres d'agriculture. Quel est l'avis de la commission spéciale ?

compléter ses missions et compétences relatives à l'animation des établissements du réseau, et de modifier en conséquence les missions des autres établissements. Quel est l'avis de la commission

aux droits de plantation de vignes, aux conventions de mise à disposition des Safer, ainsi qu'au droit de préemption dont disposent ces dernières. Pour autant, un toilettage du code rural et de la pêche maritime ne peut être envisagé qu'à droit constant. Aussi convient-il de s'assurer de l'absence d'« effets de bord » résultant d'une éventuelle abrogation des dispositions précitées.

il convient de s'assurer que ces abrogations n'ont pas d'incidence juridique. Or rien ne garantit que, en l'absence de fondement législatif, les dispositions réglementaires qui déclinent ces dispositions Dès lors, la sécurité juridique commande de conserver ces dispositions législatives, qui constituent autant de bornes légitimes à l'exercice du pouvoir réglementaire. Les professionnels eux-mêmes sont très sensibles à cet enjeu,

comprennent encore des dispositions en vigueur, dont certaines ne sont pas codifiées dans le code rural et de la pêche maritime. Dès lors, il n'est pas possible d'entreprendre un toilettage de ces lois sans risquer d'abroger des dispositions encore applicables. Compte tenu du risque posé en termes de sécurité juridique, le chantier proposé par les auteurs de cet amendement, par ailleurs tout à fait utile, nécessite, pour aboutir, une analyse plus approfondie.

La mesure proposée nécessite une étude d'impact, notamment juridique, des conséquences de l'abrogation des dispositions en cause. À la suite de la publication de la loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 tendant à améliorer la lisibilité du droit par l'abrogation de lois obsolètes, qui traitait des lois antérieures à 1940, le Sénat a entrepris un travail sur l'abrogation des lois obsolètes de la période 1941-1981. Ce travail et le véhicule législatif qui en découlera permettront, si cela est jugé opportun, d'abroger les dispositions que vous visez.

à d'anciennes décharges ou à des périmètres de protection des captages. Il y a là des espaces qui ne peuvent être consacrés à l'agriculture traditionnelle ; il importe donc que l'on puisse se saisir de ces espaces pour les destiner à d'autres usages.

cours. Nous considérons que la norme n'est pas un obstacle en soi, qu'elle est au contraire un élément de protection des populations,

un amendement d'agacement. Nous en venons donc au débat sur la protection de l'environnement. La quasi-totalité des mesures figurant dans le texte constitue une poursuite du détricotage des mesures relatives à la protection de l'environnement et à la démocratie environnementale, à l'opposé des ambitions affichées par le Gouvernement. C'est vrai ! L'affaire Lubrizol l'a montré et on l'a dit : le droit des installations classées a toute son importance, et c'est pourquoi les reculs dans ce domaine, couplés au manque de moyens pour contrôler le respect de la réglementation, font courir des risques à la population, à l'environnement, mais aussi à des activités économiques- je pense notamment à l'agriculture. Il est donc difficile de comprendre, alors que nous sommes encore en attente des résultats des investigations sur l'accident de Lubrizol, que l'on nous propose davantage de recul sur les ICPE, qui plus est dans des délais parlementaires extrêmement courts. La simplification pour les entreprises est un objectif légitime, et l'on peut parfaitement comprendre leurs besoins de clarté et de sécurité juridiques. Mais cette simplification ne passe pas nécessairement par un recul des exigences de sécurité et de participation concernant les projets.

En effet, la mesure proposée ici vise à faire bénéficier les projets en cours d'autorisation, qui ont fait l'objet d'une demande d'autorisation complète, des délais impartis aux installations existantes pour se conformer aux nouvelles prescriptions en cas de modification de la réglementation. Cette disposition conduit donc à autoriser des installations qui s'avéreront non conformes dès le jour de leur mise en fonctionnement. On peut s'interroger sur le gain de temps espéré, alors que les installations devront se conformer ultérieurement aux prescriptions. De plus, comme le souligne l'Association des maires de France, les normes ICPE font souvent, avant leur publication, l'objet de consultations avec les professionnels concernés. Ils sont donc largement informés de leur contenu, avant même la publication des textes, et ainsi en mesure d'anticiper les changements à apporter à leur projet. On peut aussi légitimement s'interroger sur les risques pour la santé et l'environnement, alors que le contrôle des ICPE existantes est actuellement très insuffisant : il a été réduit de 40 % ces dernières années. Cet article inscrit également dans la loi le principe de non-rétroactivité des nouvelles prescriptions

et ne paraît donc pas favoriser la sécurité juridique des projets. De plus, elle ne tient pas compte de l'ensemble des intérêts devant être protégés, par exemple ceux de l'agriculture ou de l'environnement, les deux étant aujourd'hui intimement liés. Pour toutes ces raisons, il apparaît nécessaire de refuser ces modifications. Merci de votre tolérance, madame la présidente ! Je considère, monsieur Labbé, que votre prochain amendement a été défendu.

puisqu'il ne s'agit que d'une application différée selon des délais définis par arrêté. Je rappelle en outre que, en cas d'enjeux importants pour la santé, la sécurité ou la salubrité publiques, il restera possible d'appliquer immédiatement les nouvelles règles à une installation en cours. L'avis est donc défavorable

à préserver le droit en vigueur applicable aux ICPE soumises au régime de l'autorisation, à savoir celles qui présentent de graves dangers ou inconvénients la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine

Cette complétude doit s'apprécier d'un point de vue formel par référence aux conditions de forme prévues par le code de l'environnement. L'aspect qualitatif des demandes est traité, après la complétude, dans le cadre de l'examen préalable du dossier

est défavorable sur l'amendement n° 150 rectifié. La problématique des prescriptions applicables aux projets en cours est identique,

Mme Céline Brulin. Par cet amendement, nous demandons la suppression de l'article L. 513-1 du code de l'environnement, qui confère des droits acquis aux entreprises en disposant que « les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration Nous nous fondons en cela précisément sur ce qui s'est passé lors de l'incendie de Lubrizol, dont je disais qu'il n'avait été tenu absolument aucun compte. Par exemple, les entrepôts de Normandie Logistique,

J'attire votre attention, ma chère collègue, sur la portée de cet amendement, qui irait bien au-delà des seuls établissements Seveso, puisqu'il impacterait l'ensemble des installations classées qui bénéficient de ce mécanisme parmi les quelque 500 000 installations existantes. Il s'agit d'un dispositif ancien du régime des ICPE qui permet de lisser l'impact dans le temps des changements de nomenclature pour les installations existantes. Nous comprenons le signal envoyé dans le cadre de l'après-Lubrizol, mais plutôt qu'une suppression brutale de ce mécanisme, il nous semble préférable de réfléchir à des mécanismes de contrôle ou de passage en revue des installations concernées en vue de vérifier l'adéquation entre leurs activités et les prescriptions auxquelles elles sont soumises. L'avis est défavorable.

environnementale sans précédent. C'est ainsi, d'abord, que les ordonnances de 2016 ont permis la mise en oeuvre d'une évaluation au cas par cas au lieu d'une évaluation systématique pour la plupart des projets. En juin 2018, un décret a réduit le périmètre des projets soumis à évaluation environnementale. Le Gouvernement a notamment décidé de soustraire les modifications des établissements Seveso à une évaluation environnementale systématique pour les soumettre à une procédure d'examen au cas relative à l'énergie et au climat ont transféré la responsabilité de la réalisation de l'évaluation environnementale au préfet lorsque le projet consiste en une modification des installations et non en une création.

existe le moindre doute sur leur engagement en faveur de notre sécurité, peut-être faudrait-il mieux répartir ces responsabilités ? L'établissement Lubrizol a, par exemple, bénéficié de ces assouplissements

l'obligation de réaliser une évaluation environnementale pour certains projets limitativement énumérés. Le code de l'environnement prévoit que, en l'absence de réponse par l'autorité chargée de cette décision dans un délai de trente-cinq jours, le projet doit être soumis à évaluation environnementale.

Or une décision implicite, d'une part, ne permet pas au maître d'ouvrage de connaître les enjeux environnementaux identifiés par l'autorité pour émettre sa décision, et, d'autre part, très difficile sa capacité à en contester le bien-fondé devant la juridiction administrative. Sans remettre en cause le mécanisme de décision implicite, le pétitionnaire doit être en mesure d'obtenir rapidement les motifs ayant conduit à cette décision. Quel

doit d'abord faire l'objet d'un recours administratif préalable. Ce recours administratif permet un dialogue entre le porteur de projet et l'autorité ayant pris la décision de soumission à évaluation environnementale, explicite ou tacite. En particulier, l'administration devra expliquer à cette occasion les motifs ayant conduit à soumettre à une évaluation

avec la réforme envisagée, la gare, les rails et les voies routières seraient donc considérés comme trois opérations distinctes, dont l'effet cumulatif des impacts ne sera donc pas évalué. Nous ne sommes donc pas favorables à cette évolution législative, et nous considérons qu'il est indispensable de prendre en compte, comme cela a été indiqué, le cumul des différents projets pour en mesurer le réel impact sur l'environnement.

qui motive le Gouvernement à agir ainsi nous semble très clair- et l'étude d'impact ne le cache pas - : il s'agit avant tout- et uniquement -de rassurer les industriels et les porteurs de projet. Là encore, l'environnement passe au second plan et nous ne pouvons malheureusement pas nous en satisfaire.

Il s'agit, une nouvelle fois, d'un amendement de suppression de deux alinéas de l'article 23, qui modifient le mécanisme d'actualisation des études d'impact de projets inscrits dans un processus d'autorisation. Aux termes de cet article, l'autorité environnementale ne revient pas sur les éléments déjà autorisés, les prescriptions nouvelles formulées ne portent que sur l'objet portent que sur l'objet de la demande concernée et, en cas de procédure d'autorisation environnementale, la consultation de l'autorité environnementale vaut à la fois pour cette procédure d'autorisation et pour l'actualisation de l'étude d'impact. Cela revient donc à affirmer le principe selon lequel l'évaluation environnementale se fait opération par opération. Or le droit européen, dans la directive Projets, interdit le « saucissonnage », c'est-à-dire le découpage par opération ou par législation de l'évaluation de l'impact d'un projet, afin de prendre en compte le cumul des différents projets et de mesurer leur réel impact sur l'environnement. Il est en effet nécessaire de revoir les prescriptions visant à protéger l'environnement de l'ensemble des activités en cas de nouveau projet, car les impacts de celui-ci se cumuleront avec ceux des installations existantes. Comme le souligne l'Association des maires de France, cet article ne semble pas prendre en compte le possible « effet domino », c'est-à-dire la propagation des effets d'un accident au-delà du strict périmètre d'une installation, qui est pourtant d'une importance capitale, comme l'a montré l'affaire Lubrizol. De même, comme l'indique France Nature Environnement, si l'on évalue séparément une gare, les rails et les voies routières attenantes, sans analyser le cumul de ces installations, comment peut-on estimer que l'on prend en compte l'impact réel d'un projet ? Enfin, les incohérences entre cet article et le droit européen peuvent également fragiliser les projets, qui pourraient être remis en cause pour non-conformité. Cela va, encore une fois, à l'inverse de la recherche de simplification et de sécurité juridique. Cet article constitue un recul important, et c'est pourquoi nous aussi souhaitons sa suppression.

pour ma part favorable à ce que l'on rende le droit plus lisible pour les porteurs de projet. Il est nécessaire de préciser que l'actualisation d'une étude d'impact et le nouvel examen par l'autorité environnementale ne font pas peser de risque sur les autorisations déjà données. Il s'agit bien de rassurer les industriels et de privilégier plutôt l'implantation de nouveaux projets sur des zones industrielles déjà existantes. L'avis est donc défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Dès 2017, dans le cadre de la ratification des ordonnances, nous avions proposé de revenir sur la frontière trop stricte entre « cas par cas » et évaluation automatique. la Cour de justice de l'Union européenne, la marge d'appréciation laissée aux États membres pour fixer des seuils trouve sa limite dans l'obligation qu'un projet fasse l'objet d'une étude d'impact, dès lors qu'il est susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement, et, en outre, la fixation de seuils ne permet jamais de prendre en considération le critère de cumul d'effets avec ceux d'autres projets, ce cumul pouvant s'analyser seulement. Ces considérations avaient conduit d'ailleurs le groupe de travail sur la modernisation du droit de l'environnement, dirigé par Jacques Vernier, à proposer l'introduction d'une « clause-filet » ouvrant la possibilité de soumettre à évaluation environnementale un projet que l'on pourrait qualifier de « petit », non visé par le régime de l'examen au cas par cas, mais situé dans un milieu sensible ou fragile ; tel est manifestement le cas de la prévention des risques industriels, notamment ceux liés aux effets « domino » ou « cocktail ». L'objet de cet amendement, que nous présentons chaque fois que nous le pouvons parce qu'il nous semble extrêmement pertinent, est donc de mettre la législation en conformité avec le droit de l'Union européenne, pour lequel les seuils ne sont qu'indicatifs, et d'ouvrir la possibilité au pouvoir exécutif de mettre en oeuvre rapidement cette fameuse clause-filet. Quel

afin de pouvoir, si c'est justifié, les soumettre à évaluation environnementale. Il prévoit ainsi que sont soumis à évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement en fonction de critères ou » de seuils définis par décret, et non pas en fonction de critères « et » de seuils. De cette manière, l'autorité compétente pourrait saisir l'autorité environnementale afin d'examiner s'il est nécessaire de soumettre un petit projet à évaluation environnementale. L'idée est de dire que ce n'est pas parce qu'un projet est « petit » en taille qu'il n'a pas d'impact sur l'environnement. La France a fait le choix de fixer des seuils pour déterminer les projets devant faire l'objet d'une évaluation environnementale, systématique ou au cas par cas. La directive européenne nous le permettait. Nous avons usé de cette possibilité. La mesure proposée serait potentiellement très lourde pour certains petits projets, agricoles notamment. N'importe quel permis de construire pourrait potentiellement être concerné. Je pense que l'on créerait ainsi

2019. Quel est l'avis du Gouvernement ? La nomenclature actuelle de l'évaluation environnementale permet déjà de distinguer les seuils et critères selon les types de projets et les milieux dans lesquels ils s'insèrent.

le premier signataire. Il a pour objectif de garantir que tout projet ayant des incidences notables sur l'environnement fasse l'objet d'une évaluation environnementale, de la directive Projets, et à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui estime qu'un projet, de dimension même réduite, peut avoir de telles incidences

que la législation française n'est pas conforme à la directive européenne en ce qu'elle exclut des projets ayant des incidences sur l'environnement de toute évaluation et fixe des seuils d'exemption inadaptés. Le présent amendement vise donc à se conformer au droit européen et reprend la proposition du

et/ou critères retenus pour l'application de cette obligation. Il permet également à l'autorité compétente, ou au maître d'ouvrage, de saisir l'autorité environnementale afin de procéder à un examen au cas par cas, et donc de sécuriser juridiquement les projets.

Le présent amendement vise à garantir l'indépendance de l'autorité environnementale, à l'instar de ce que prévoient les dispositions en matière de plans et de programmes, en la dissociant de l'autorité compétente en matière d'autorisation. Il vise à prévenir les contentieux en la matière et donc à sécuriser les projets. Il s'agit également de

et que les moyens sont insuffisants pour l'examen des autres évaluations pertinentes. L'absence de clause de rattrapage constitue une régression dans l'application du principe de prévention de prévention des atteintes à l'environnement et un recul en matière d'acceptabilité des projets. Elle représente donc un risque d'insécurité juridique pour les porteurs de projet. Or le Conseil d'État, dans sa décision du 8 décembre 2017, a confirmé confirmé qu'« une réglementation exemptant de toute évaluation environnementale un type de projets antérieurement soumis à l'obligation d'évaluation environnementale après un examen au cas par cas n'est conforme au principe de non-régression de la protection de l'environnement que si ce type de projets, eu égard à sa nature, à ses dimensions et à sa localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la

en prenant en compte des éléments contenus dans ce rapport. Je pense notamment à la nécessité d'acculturer les industriels aux enjeux environnementaux et à la réglementation, ainsi qu'à l'importance de donner véritablement davantage de poids à la consultation du public, ce que certains qualifient de « redevabilité », c'est-à-dire la justification de la prise en compte des avis des citoyens et de l'autorité environnementale. Je n'y reviendrai pas longuement, mais ce qu'a aussi montré l'accident industriel de Lubrizol, c'est la nécessité de tenir compte des inquiétudes légitimes et des avis des populations, voire de construire avec elles un certain nombre de réponses. Le rapport

citer la présentation de l'action 9 sur l'accélération des procédures, et ce regret, formulé sur la question plus large de la consultation du public : « La mission constate et regrette une prise en compte trop limitée de l'avis des citoyens lors du processus d'enquête publique. Pour y remédier et sans aller vers des solutions contraignantes, il conviendrait de concevoir et d'envisager des mécanismes plus innovants pour associer davantage les citoyens. » Nous voulons pour notre part, aller en ce sens, et respecter l'esprit de la convention d'Aarhus en passant d'une simple

de deux manières : premièrement, en lui permettant de réagir à la réponse écrite du maître d'ouvrage à son avis en formulant un avis complémentaire à la demande du commissaire enquêteur ; deuxièmement, en obligeant l'autorité chargée de l'autorisation du projet à justifier la non-prise de mesures en cas d'incidences résiduelles

est que l'autorité chargée de décider de cette soumission ne soit pas la même que celle chargée de donner l'autorisation. La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable avait déjà souligné, à l'occasion de l'examen de la loi relative que cette solution continuait de poser problème, dans la mesure où elle permettait à un préfet d'être à la fois celui qui décide si un projet doit faire ou non l'objet d'une évaluation environnementale et celui qui est compétent pour autoriser ce projet. Elle avait d'ailleurs proposé que l'autorité désignée pour assurer l'examen au cas par cas des projets dispose également d'une autonomie fonctionnelle par rapport à l'autorité compétente pour autoriser le projet,

au climat, une disposition qui permet de trouver un juste équilibre entre autorité environnementale et autorité chargée de l'examen du projet au cas par cas.

En effet, nous constatons souvent sur le terrain que l'administration laisse fréquemment les entrepreneurs sans réponse, alors qu'ils ont déjà engagé des frais et mobilisé des ressources pour lancer de nouveaux projets. Ainsi, dans le Nord, un entrepreneur a demandé à l'autorité compétente s'il devait engager une étude d'impact. Sans réponse de l'État pendant un an, il a décidé d'engager les travaux, et c'est seulement à ce moment-là que l'administration s'est réveillée pour le sanctionner

Ma première remarque concerne la lisibilité du dispositif proposé par l'amendement : je ne suis pas sûre de comprendre ce que voudrait dire une « acceptation » dans le cas d'une procédure de cas par cas. En effet, l'autorité compétente doit décider si, oui ou non, un projet doit être soumis à évaluation environnementale. Que voudrait donc dire un silence valant acceptation ? Le projet serait-il soumis à évaluation environnementale en cas de silence ? Deuxième remarque, je rappelle que ce qui justifie la règle du refus implicite en cas d'absence de réponse correspond à des enjeux de sécurité publique et de protection de l'environnement. Enfin, l'autorité environnementale dispose d'un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du formulaire complet pour informer, par décision motivée, le porteur de projet de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. La préoccupation exposée dans l'amendement étant en partie satisfaite,

Il fait donc l'objet d'une étude d'impact systématique dès que le débit de l'appareil projeté dépasse les 1 500 personnes à l'heure, ce qui est le cas de tous les téléportés créés Néanmoins, le remplacement d'une remontée mécanique s'accompagne bien souvent d'une diminution du nombre de pylônes, compte tenu des progrès de la technique, et n'entraîne pas d'impact significatif supplémentaire sur une zone déjà aménagée.

(DHUP) et de France Nature Environnement. Pourtant, la modification n'a pas été prise en compte dans les textes. Aussi, cet amendement a pour objet de permettre une dispense d'étude d'impact systématique lors du remplacement d'une remontée mécanique. Quel est l'avis de la commission Les projets de remontées mécaniques transportant plus de 1 500 personnes sont aujourd'hui soumis à évaluation environnementale systématique. Cet amendement vise à déroger à cette systématicité en prévoyant la possibilité de dispenser le maître d'ouvrage d'une étude d'impact pour les projets de remplacement de remontées mécaniques ou téléphériques. Tout d'abord, le champ des projets soumis à étude d'impact est de nature réglementaire : il est défini dans un tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, à la rubrique 43 pour les projets de remontées mécaniques et de téléphériques. En outre, il est prévu que les travaux de remplacement à l'identique des remontées mécaniques, qui sont assimilables à des travaux de maintenance ou de grosses réparations, sont exemptés de l'obligation de soumission à évaluation environnementale. En revanche, les travaux de remplacement qui ont pour effet d'augmenter la capacité de transport de la remontée mécanique peuvent être considérés comme des extensions et, dès lors, soumis à examen au cas par cas dans la grande majorité des cas et, pour les augmentations les plus importantes, à évaluation environnementale systématique.

? Compte tenu du métier que j'exerçais précédemment, je me contenterai de lire la fiche de banc préparée par les ministres compétents. En premier lieu, je souhaite rappeler que le champ de l'évaluation environnementale relevant du domaine réglementaire, il ne revient pas à la loi de préciser les exemptions en la matière. En second lieu, sur le fond, les travaux de remplacement à l'identique des remontées mécaniques sont déjà exemptés d'évaluation environnementale, en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans la mesure où ils sont assimilables à des travaux de maintenance ou de grosses réparations. Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale. » Le droit actuel permet donc déjà de répondre pleinement au souhait des auteurs de cet amendement. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Cet amendement concerne les études d'impact environnemental. Sans justification par rapport au droit européen, cette exigence générale d'une étude d'incidence pour tout projet qui ne fait pas l'objet d'une évaluation environnementale constitue une surtransposition. Si l'obligation d'une étude d'incidence peut se justifier, sa généralisation à tous les cas pour lesquels il n'y a pas obligation d'évaluation environnementale semble excessive et injustifiée. En effet, ce n'est qu'au terme d'un examen au cas par cas que le porteur de projet saura, dans le cas où cet examen conclura à l'absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale, qu'il doit faire une étude d'incidence environnementale. Cela conduit le pétitionnaire à supporter deux fois une procédure sans aucune justification légale, tant au niveau européen que national. Quel Supprimer ici l'obligation d'une étude d'incidence, dans une autorisation qualifiée d'environnementale, ne permettrait pas à l'autorité décisionnaire- le préfet -de prendre la décision d'autorisation ou de refus en toute connaissance de cause. En effet, l'absence d'étude d'impact ne signifie pas que le projet n'a absolument aucune incidence sur l'environnement, et ce d'autant que les seuils relatifs à l'étude d'impact ont été relevés ces dernières années. Un projet qui n'est pas soumis à évaluation environnementale n'est pas pour autant dénué de tout impact sur l'environnement. L'avis est donc défavorable. donc défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ? Je tiens à préciser que le porteur de projet commencera par renseigner un formulaire « cas par cas » comportant les informations nécessaires à l'autorité compétente pour décider si l'étude d'impact est requise. Ce n'est que lorsqu'il est dispensé d'étude d'impact

Je souhaitais prendre la parole sur l'article 24 pour m'exprimer plus largement sur les dispositions du présent projet de loi relatives au régime des installations classées pour la protection de l'environnement. Comme vous le savez, madame la secrétaire d'État, le Sénat a créé, à la demande de l'ensemble des présidents de groupes et de commissions, une commission d'enquête pour analyser la gestion des conséquences de l'incendie de l'usine Lubrizol du 26 septembre 2019, et en tirer des enseignements pour l'avenir. J'ai l'honneur d'en être l'un des vice-présidents. Mon objectif est, à cet instant, non pas de m'exprimer au nom de la commission d'enquête, qui présentera ses conclusions d'ici au début du mois d'avril, mais de vous faire part, à titre personnel, de certaines réserves par rapport à ce projet de loi. Je regrette vivement le signal qu'envoie le Gouvernement en proposant des mesures guidées par le seul souci de simplifier la vie des industriels. Ces propositions proviennent d'un rapport remis au Gouvernement par notre collègue député Guillaume Kasbarian le 23 septembre 2019, c'est-à-dire trois jours avant l'accident de l'usine Lubrizol. Ce rapport était guidé par le souci d'alléger les contraintes administratives des entreprises. À mon sens, le contexte et les attentes de la population ont profondément changé depuis : c'est peu dire que la population de Rouen a été très mécontente du manque d'information sur les risques industriels liés, notamment, à la présence d'une industrie chimique puissante au sein même de l'agglomération.

Traiter les procédures de consultation du public comme un fardeau ne contribuera pas à améliorer l'acceptabilité des activités industrielles. Au contraire, les réactions à l'accident de l'usine Lubrizol témoignent d'une véritable crise de confiance dans nos territoires à l'égard de la maîtrise des risques industriels. Les mesures proposées ne vont pas dans le bon sens. J'observe d'ailleurs qu'elles entrent en contradiction avec les propos tenus devant notre commission d'enquête par plusieurs ministres, qui ont déploré le manque de culture du risque dans notre pays. En outre, sur la forme, je m'étonne que le Gouvernement propose dès à présent des dispositions sur ce sujet, alors que plusieurs prises de parole avaient laissé entendre que l'exécutif attendrait les conclusions des travaux des deux assemblées avant de proposer des évolutions. Force est de constater que cette méthode n'a pas été respectée. Permettez-moi donc d'espérer qu'à l'avenir le Gouvernement prêtera plus d'attention aux travaux de contrôle du Parlement et saura mieux mettre en cohérence ses actes avec ses paroles.

avait d'ailleurs invité le Gouvernement à préciser dans l'étude d'impact les cas où il envisageait de conserver une information systématique des commissions dans le cadre de dispositions réglementaires.

Comme le précise l'étude d'impact, « dans les cas où le préfet choisira [ ...] de ne pas consulter le Coderst, cela contribuera à raccourcir de plusieurs semaines le délai total d'autorisation d'une implantation industrielle, avec des gains indirects non négligeables sur l'économie du projet on oppose l'économie et l'environnement, alors qu'au contraire, dans notre monde moderne, face aux enjeux et aux risques qui pèsent sur nous, il faudrait

une urgence sociale, une urgence environnementale et une urgence démocratique. Là encore, on amoindrit les procédures de consultation et de concertation, alors que nos concitoyens

à l'encontre d'une plus grande association des citoyens aux décisions environnementales. Nous sommes à l'opposé d'une réponse au désir de participation exprimé par la population lors du grand débat. Cette concertation via les Coderst est très utile, car elle permet à différents acteurs locaux de souligner des enjeux dont l'administration n'a pas nécessairement connaissance et ainsi d'éclairer les décisions du préfet. Le Coderst est la seule instance départementale dans laquelle des représentants d'associations de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement notamment, ou encore des médecins, se réunissent pour évaluer les risques d'un projet pour la santé et l'environnement. Il est d'autant plus dommageable de se priver de cette concertation que le gain de temps attendu de cette réforme pour les porteurs de projet est très modéré, de l'ordre de deux semaines, de l'aveu même de la commission spéciale dans son rapport. La seule ambition du texte semble donc bien être l'accélération des projets. Rien ne semble aller dans le sens de la recherche d'un juste équilibre entre le développement industriel, qui est- je le rappelle -nécessaire, et la protection de l'environnement et des riverains. De plus, cet article semble remettre en cause le rôle du Coderst, auquel de moins en moins de dossiers sont présentés, du fait du basculement de nombreux ICPE vers le régime de l'enregistrement. Il s'agit donc d'un recul majeur pour la démocratie environnementale qui pourrait, par ailleurs, donner lieu à des contentieux- certains sont d'ailleurs déjà en cours et la situation risque de s'aggraver. Encore une fois, ces mesures

Ces amendements identiques visent à supprimer l'article rendant facultative la consultation du Coderst ou, le cas échéant, de la CDNPS. La commission spéciale a considéré qu'il s'agissait d'une évolution permettant une simplification proportionnée, offrant un gain en termes de délai pour la procédure d'enregistrement, de l'ordre de trois à quatre semaines. Le préfet gardera bien sûr la possibilité de consulter la commission compétente, en fonction des enjeux du projet et de la situation locale. Le représentant de l'État sait apprécier la sensibilité du projet, car, à la suite de la réforme, 70 % des projets soumis à autorisation continuent de faire l'objet d'une consultation de la commission départementale. L'avis est défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ?

que c'est parce que l'on a basculé un certain nombre d'installations soumises à enregistrement qu'il y aurait moins de dossiers devant les Coderst. Ce serait plutôt le contraire ! La réalité, c'est qu'il y a moins de dossiers d'extension et d'installation de nouveaux sites,

prescriptions standard, seront obligatoirement soumis au Coderst. En revanche, si le préfet durcit les prescriptions

précédemment. L'article 24 supprime la consultation systématique du Coderst ou de la CDNPS pour des projets relevant notamment des régimes d'enregistrement. Sans revenir sur le caractère facultatif d'une consultation de ces commissions et conseils pour les demandes d'autorisation environnementale soumises à évaluation environnementale, il est proposé d'ouvrir un droit d'option pour le porteur de projet. Il semble

en l'absence de consultation, la commission est en tout état de cause informée. Surtout, le porteur de projet a déjà la possibilité de solliciter l'administration en vue de la consultation de la commission. Il n'y a aucune raison que le préfet ne donne pas suite

de cet article, nous vous demandons d'entendre la Compagnie nationale des commissaires enquêteurs, qui en demande la suppression. En effet, la participation du public est un élément incontournable de l'élaboration de la décision ; elle est nécessaire à l'amélioration de la qualité des projets et donc à leur acceptabilité par nos concitoyens. Vouloir réduire cette mesure à une simple consultation du public par voie électronique

d'ailleurs pas davantage de garanties, puisqu'elle n'exclura absolument pas les recours contentieux lourds de conséquences, notamment financières, pour les porteurs de projet. de projet. Cette procédure de consultation fait douter de son efficacité en termes de restitution des observations. Lorsque des observations sont déposées, il est constaté qu'au final l'arrêté préfectoral ne fait état

Voici ce qu'elle m'a écrit : « Je m'adresse à vous aujourd'hui en votre qualité de sénateur au sujet du projet de loi ASAP. Le texte proposé vise en son article 25 à " permettre au préfet de choisir entre une consultation électronique du public ou une enquête publique pour certains projets soumis à autorisation ne nécessitant ne nécessitant pas d'étude d'impact environnemental ". « Outre le fait que le respect de la convention d'Aarhus, ratifiée par la France, est mis à mal par le renforcement des pouvoirs régaliens et discrétionnaires du préfet, la disparition de l'enquête publique aurait de nombreux effets négatifs, notamment écarter toute possibilité d'expression orale des citoyens et des associations telle qu'elle se pratique lors des permanences des commissaires enquêteurs et durant toute la consultation tout moyen de dialogue, d'approfondissement et de saisie d'observations pertinentes en résultant, car impossible par la seule approche dématérialisée pour le maître d'ouvrage, faire disparaître la possibilité, prévue par la procédure d'enquête, de répondre aux observations du public ; supprimer l'opportunité de disposer d'un avis indépendant et éclairé, permettant d'améliorer la qualité de la décision administrative et renforçant sa légitimité. « Par ailleurs, cette recherche de réduction des délais par la suppression pure et simple de l'enquête publique,

qui contrevient au principe de la Charte de la participation du public [ ...] qui dans son préambule précise que " la participation du public est un élément incontournable de l'élaboration de la décision, nécessaire à l'amélioration de sa qualité et de sa légitimité " . » Je suis

qui vise à remplacer les procédures actuelles par une simple consultation du public par voie électronique. Pour ne pas allonger inutilement les débats, souligner que le Conseil d'État est lui-même extrêmement réservé sur cet article, ce qui donne un argument supplémentaire, me semble-t-il, pour en plaider la suppression.

enjeux locaux. Pour ces projets, le maintien d'une enquête publique semble nécessaire. Cette procédure est en effet bien plus complète qu'une simple participation par voie électronique. écarte du projet la partie du public qui n'est pas familière avec l'informatique. Conduite par un commissaire enquêteur indépendant et impartial, à la fois garant de la qualité de la participation et chargé de formuler un avis, l'enquête publique permet une véritable information du public et des échanges avec les citoyens. citoyens. De plus, je le redis, on constate que les procédures électroniques, dans un contexte de fracture numérique, rendent difficile la participation de certains citoyens. Réduire ainsi le champ des enquêtes publiques

En effet, il paraît de bon sens de laisser la possibilité au préfet d'adapter la procédure de consultation du public pour les projets dénués d'impact environnemental important. Aujourd'hui, tous les projets soumis à autorisation environnementale doivent faire l'objet d'une enquête publique, même ceux qui ne sont pas soumis à évaluation environnementale, c'est-à-dire qui n'ont pas d'incidence notable sur l'environnement. Or, comme nous l'ont expliqué les services que nous avons entendus, les retours sur les enquêtes publiques de projets non soumis à évaluation environnementale sont d'ampleur très variable : concrètement, sur certains dossiers, personne ne se déplace. On parle d'autorisations de projets tels que de grandes stations-service ou de gros pressings. Cet article permet au préfet d'apprécier si une participation par voie électronique n'est pas suffisante. Cette mesure,

feront de toute façon l'objet d'enquêtes publiques. Pour ceux qui ne sont pas soumis à l'évaluation environnementale, on distingue ceux qui présentent de forts enjeux locaux, pour lesquels le préfet conservera l'enquête publique, de ceux qui n'induisent pas de tels enjeux, pour lesquels le préfet opérera

Vous aviez droit à une erreur dans la matinée, vous l'avez faite ! On entend trop cela. N'oublions pas que l'environnement et la biodiversité sont en péril ! Il ne faut pas tout mélanger.

la secrétaire d'État. Je lis le début de l'exposé des motifs du projet de loi : « Le grand débat national a mis en lumière les attentes majeures des Français [ ...] Les Français ont à cette occasion exprimé une forte demande de services publics, plus proches, plus lisibles, adaptés aux usagers et accessibles dans tous les territoires. Ils ont insisté sur un besoin de proximité [ ...] » Je ne vois pas en quoi le fait de passer par une consultation numérique au lieu d'aller en mairie et de rencontrer les gens répond à cet exposé des motifs et à ce besoin de proximité.

sort meilleur ... Cet amendement vise à permettre au préfet de recourir à l'enquête publique lorsqu'un projet faisant l'objet d'une procédure d'autorisation, mais n'étant pas soumis à évaluation environnementale, est susceptible d'avoir un impact sur la santé humaine. Les enjeux socioéconomiques peuvent être pris en considération dans ce cadre, mais l'impact sur la santé humaine nous semble constituer un intérêt au moins aussi fondamental à protéger. Compte tenu de la technicité de certains dossiers, l'intervention d'un commissaire enquêteur indépendant permettra de mener une consultation du public qui soit plus objective et éclairante que la simple participation par voie électronique.

Le domaine public maritime naturel est l'un des plus vastes domaines de l'État. Les préfets de département ont la charge d'administrer ce domaine en veillant à concilier ses différents usages et en intégrant au mieux les enjeux environnementaux. Les préfets ont été nombreux à mettre en évidence le besoin de simplifier certaines procédures, notamment celles qui sont liées à la délimitation ou aux concessions d'utilisation. Cet amendement vise à répondre à ces attentes, également relayées, pour ce qui concerne les concessions, par les collectivités locales qui administrent les ouvrages de protection de la population face aux risques littoraux. auteurs d'un rapport récent sur la mise en oeuvre des plans d'action et de prévention des inondations appellent de leurs voeux une mise en oeuvre rapide de la mesure de simplification relative aux concessions. Cet amendement tend également à sécuriser les procédures de création de servitudes de passage de piétons sur le littoral ; l'objectif est de renvoyer ces créations à la procédure d'enquête publique prévue par le code des relations entre le public et l'administration, moins lourde que la procédure actuelle, rattachée au code de l'expropriation. Environ 5 800 kilomètres linéaires de sentiers du littoral sont ouverts en 2019 sur l'ensemble des côtes françaises, dont 1 530 kilomètres au titre de la servitude de passage des piétons. Avec cette mesure, le Gouvernement entend consolider la procédure de création de plus de 1 000 kilomètres linéaires de sentiers, qui sont encore à l'étude, afin de garantir l'accès des Français au rivage de la mer. a donc pour objet d'introduire plusieurs simplifications, qui correspondent aux attentes des parties prenantes et qui seront bénéfiques à la gestion du domaine public maritime.

cet article, même si je vois bien qu'il concerne des cas assez particuliers. Le fait de permettre, en gros, à des industriels de commencer des travaux

mesure] se traduit par une troisième décision administrative du préfet ». En outre, cela nuira à la lisibilité des procédures pour nos concitoyens, qui pourront voir des travaux se lancer

cela ne sera possible qu'à condition que les deux consultations du public aient été dissociées et que le permis de construire ait donné lieu à une consultation du public mentionnant le démarrage anticipé.

Je redis les conditions d'application de cet article : information préalable du public, démarches effectuées aux frais et risques du demandeur, permis de construire délivré- il y a donc évidemment une autorisation

pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur un nouveau bâtiment destiné à accueillir des activités équestres. Pour des raisons topographiques et d'accès au bâtiment, la communauté a dû déplacer de 120 mètres, sur le même site, l'emprise du bâtiment.

une nouvelle instruction par les services de l'État ; c'est une forme de suradministration ... Résultat : le bâtiment a été inauguré le 1 février dernier sans toiture photovoltaïque, alors que le point de raccordement et les caractéristiques techniques du projet n'ont guère été modifiés.

Si nous souhaitons concrétiser nos ambitions en matière de production d'énergies renouvelables, le bon sens doit revenir dans nos pratiques administratives, comme l'indique l'intitulé de ce texte, « accélération et simplification de l'action publique ».

Si l'objectif de cet amendement est louable, puisqu'il vise à mieux articuler différentes autorisations issues du code de l'urbanisme et du code de l'énergie, il pose plusieurs difficultés. D'abord, il tend à priver de leurs attributions non seulement les maires, puisqu'une autorisation modifiant la construction au titre du code de l'urbanisme n'aurait plus nécessairement d'incidence sur l'autorisation permettant l'exploitation au titre du code de l'énergie, mais encore les préfets, qui ne disposeraient plus d'un pouvoir d'appréciation dans la délivrance de l'autorisation d'exploitation prévue par ce second code. Ensuite, l'amendement n° 48 rectifié n'est pas borné, de sorte que l'autorisation demeurerait acquise sans contrainte de temps. Enfin, Enfin, le dispositif aurait sans doute peu d'applications concrètes puisqu'il pose comme condition que les caractéristiques techniques de l'installation soient identiques. Or la modification de la construction a très souvent un effet sur les caractéristiques de l'installation.

La localisation d'une installation produisant des énergies renouvelables est un élément fondamental dans la décision d'autoriser ou non un projet, notamment pour déterminer les impacts sur l'environnement ou sur le voisinage. L'article L. 311-6 du code de l'énergie prévoit déjà que les installations dont la puissance est inférieure à un seuil défini par décret sont réputées autorisées. Par conséquent, pour celles-ci, aucune démarche n'est à accomplir.

entraîne la soumission au régime de l'autorisation environnementale et permet donc une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux. L'article 23 de la loi OFB, issu justement

que les projets en cours, dont la demande a été déposée avant la publication de la loi, ne soient pas concernés par cette nouvelle définition des zones humides. On peut comprendre que l'on recherche la sécurité juridique de ces projets. Mais, si cet objectif est louable, on sait les zones humides constituent un enjeu majeur en termes de biodiversité et fournissent des services environnementaux essentiels en termes de protection des ressources en eau et de captation du carbone. Il est important, au regard de ces enjeux, que la nouvelle définition des zones humides s'applique également aux projets en cours. Il convient donc de soutenir cet amendement de suppression pour éviter la destruction d'un nombre pour l'instant inconnu, mais non négligeable, de milieux humides. À cet égard, je salue la position du Gouvernement sur l'amendement.